La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur la mixité sociale à l'école, à la demande du groupe socialiste, écologiste et républicain. Et la parole et tout d'abord à l'orateur du groupe, qui a demandé ce débat donc c'est madame Sylvie Robert pour le groupe socialiste, écologiste républicain qui va s'exprimer pour huit minutes. Bien monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les établissements scolaires français sont touchés par un phénomène puissant de ségrégation sociale qualifié je cite de bombe à retardement pour la société française par Nathalie Mons ancienne présidente. Du Conseil national d'évaluation du système d'évaluation scolaire ce constat dressé en 2015 n'est malheureusement pas nouveau depuis près de 20 ans. Les études se succèdent et souligne que les indicateurs de mixité sociale à l'école ne s'améliore pas pire la dernière étude Pisa de 2018 démontré à quel point le système scolaire français devenait gravement inégalitaire sous le poids des déterminismes sociaux avec Israël et le Luxembourg, la France est le pays de l'OCDE où l'origine sociale des parents influencent le plus le parcours scolaire. Or nous ne pouvons nous satisfaire d'une telle représentation à moins d'estimer que le retour à une société de classe figé est un projet politique d'avenir. La récente publication des indices de position sociale IPS des collèges et des lycées a jeté une lumière crue sur le déclin de la mixité sociale dans notre système scolaire. Ainsi, sur les 100 premiers lycées ayant des IPS les plus élevés, 82 sont des établissements privés sous contrat. Cette véritable saignée du secteur public est accompagnée d'un double mouvement profond. D'une part de terribles disparités au sein même du système scolaire, notamment entre la filière professionnelle et c'est le général et technologique. La moyenne des IPS des lycées généraux et technologiques, privé et public confondus, est de 114 21 quand celle des lycées professionnels n'est que de 87,5, presque 30 points d'écart. Nous rendons-nous compte mes chers collègues ce que dévoile ses chiffres les sociologues de l'éducation ont un terme pour désigner cette dichotomie au sein du système scolaire le tri social. D'autre part les inégalités territoriales très fortes sont à l'oeuvre certaines académies concentrant la plupart des établissements à faible ou fort IPS, ce qui témoigne en filigrane de l'importance des politiques de logement et d'aménagement du territoire, mais j'y reviendrai. Désormais, la question qui nous est adressé, en tant que décideur politique est de savoir si nous voulons réellement renforcer la mixité sociale à l'école facteur déterminant de réussite scolaire, singulièrement pour les élèves défavorisés ou si à l'inverse, nous estimons qu'elle est un sujet mineur voire une fatalité. Monsieur le Ministre, d'après vos propos vous avez clairement opté en faveur de la première hypothèse et le groupe socialiste, écologiste et républicain s'en réjouit. En effet, nous sommes convaincus que l'absence de mixité scolaire à l'école n'est ni acceptable ni soutenable aucunement acceptable car elle induit une conception séparatiste de notre société, ainsi qu'une indifférence généralisée aux inégalités qu'elle engendre. Aucunement soutenable, car elle gangrène l'idéal cardinal d'égalité des chances au fondement de notre pacte républicain. Si l'école ne permet plus d'assurer la mobilité sociale, c'est l'ensemble de notre édifice sociétal et démocratique qui est en danger. Pourtant, 2000 depuis 2013 et la loi d'orientation et de programmation pour une refondation de l'école, la mixité sociale est un objectif du service public de l'éducation qui doit, je cite, veiller à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements, tout en contribuant à l'égalité des chances et à la lutte contre les inégalités sociales et et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Dès lors comment combler l'écart entre la théorie et la pratique. Ou si vous préférez, entre la loi et la réalité constatée. Le gouvernement socialiste en collaboration avec les collectivités territoriales volontaires s'est attelé à apporter une première réponse en 2016 suite au plan mixité Scola social dans les collèges initiée par la ministre de l'Éducation nationale. 17 départements ont lancé des expérimentations pour lutter contre la ségrégation sociale dans le secondaire. À cet égard. Le plan mis en oeuvre par le département de la Haute-Garonne présente des résultats remarquables et une conclusion incontestable peut en être tiré. La mixité sociale permet aux élèves défavorisés de mieux réussir scolairement sans pour autant faire baisser, bien sûr, la réussite des élèves les plus favorisés, en pratique elle établit donc un système gagnant gagnant aussi le plan Haute-Garonne elle témoigne que plusieurs ingrédients sont indispensables pour garantir le succès de telles initiatives. Le temps de la concertation cher Émilienne en particulier avec les parents La co-construction avec la communauté éducative faire évoluer positivement le projet et assure son acceptabilité globale des moyens budgétaires sont impératifs, lesquels peuvent porter sur des politiques publiques connexes. Je pense à la mobilité, notamment au bus scolaire par exemple, et bien sûr l'appui du ministère de l'Éducation nationale, y compris financier est primordial. Par conséquent monsieur le ministre allez-vous soutenir plus massivement ses expérimentations territoriale qui ont vraiment un impact éducatif et social évident et êtes-vous prêt à dégager des moyens pour accompagner ces collectivités territoriales qui seraient volontaires. Cette question est d'autant plus légitime que nous savons vos chantiers nombreux rémunération des professeurs généralisation de l'école du futur même si je n'entends plus parler beaucoup de ce terme-là concrètement de quel budget disposez vous disposez-vous pour compte. Accroître la mixité sociale à l'école, j'insiste, mais ce point est essentiel car au-delà des adaptations organisationnelles, que vous proposerez il déterminera la portée réelle aussi de votre action. Car sans ressources budgétaires adéquates point de plan ambitieux en matière de mixité sociale. Autre problématique abordée en préambule mon intervention. La participation du privé sous contrat à l'objectif de mixité sociale au regard de l'ampleur du phénomène de ségrégation sociale qui a fait que le système scolaire est-il encore possible de fermer les yeux et de laisser faire. C'est la question que je vous pose, que je nous pose collectivement, mes chers collègues, la liberté de recrutement du privé est-elle négociable aujourd'hui. J'ajouterais qu'en France, sauf erreur de ma part nulle liberté n'est absolue. Si bien que, comme toute liberté, la liberté de recrutement peut être encadré dans la mesure où elle constitue un enjeu décisif pour améliorer la mixité sociale à l'école et la réussite de tous les élèves ce sont l'efficacité et la crédibilité de notre politique éducative publics qui sont en jeu, en finançant les établissements privés sous contrat à hauteur de 73%, sans contrepartie en matière de mixité sociale, l'État ne participe-t-il pas de l'éviction du public vers le privé et l'État ne fera la-t-il pas finalement ses propres écoles publiques. Alors Monsieur le Ministre, allez-vous par exemple moduler peut-être les dotations des établissements privés sous contrat en fonction de leur action ou inaction en matière de mixité, êtes-vous favorable à cette conditionnalité comme vous le constatez, cette proposition ne vise nullement à punir les écoles privées mais bien à faire en sorte qu'elle concourt à cet objectif de Miss quitter social et scolaire plus globalement en fait que comprendra le protocole d'accord que vous envisagez. Enfin, la mixité sociale des établissements scolaires dépendent des politiques de logement et d'aménagement du territoire. Avez-vous entrepris un travail interministériel avec vos collèges du ministère de la transition écologique de la cohésion des territoires et aussi bien sûr en lien avec les collectivités territoriales. Et si la réponse est positive sur quelle conclusion peut-être pourraient-ils aboutir. Alors, mes chers collègues après le combat en faveur de l'égal accès aux études qui fut celui du XXe siècle schématiquement celui en faveur de l'égalité des chances demeure entier et probablement peut-être plus intense, encore que dans les années 80. Car si l'école ne peut pas tout, la promesse méritocratique qui lui est attachée doit impérativement être rehaussée. Ce qui implique de s'assurer que les conditions de sa réalisation pour tous soit réunies par se passer de la partialité des chances à une régate réelle égalité des chances oblige à un volontarisme politique très fort et affirmé afin de brider briser les ghettos sociaux et scolaires, sous peine de basculer vers une société purement endogame ou même dans un gouffre démocratique. Je vous remercie. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les madame la sénatrice Robert avec votre groupe vous avez souhaité inscrire à l'ordre du jour du Sénat. Un débat sur la mixité sociale au sein des établissements scolaires. Je vous en remercie puisque j'ai placé dès mon arrivée au ministère ce sujet comme une priorité de mon action et je vous en remercie parce que ce sujet nécessite la mobilisation, l'engagement et la la persévérance de tous, en particulier les collectivités locales que vous représentez au sein de cette assemblée. La mixité sociale et scolaire dans les écoles et les établissements est une des conditions de la réussite de chaque élève. La diversité des parcours familiaux, la multiplicité des origines sociales leurs mélanges et leurs interactions sont une force et non une faiblesse pour l'école, l'école doit porter, c'est son rôle. Une vision émancipatrice de son action auprès des élèves. Elle doit lutter contre les déterminismes de naissance d'origine ou de genre, elle doit permettre à chaque enfant. D'étendre ses ambitions au delà de ce à quoi son environnement le restreint, voire le contraint. Malgré les efforts engagés depuis plusieurs années, la France est en effet un des pays de l'OCDE où les déterminismes sociaux pèsent le plus sur la réussite scolaire des élèves au delà même de la réussite scolaire les phénomènes ségrégative prive la société de talent bride les ambitions décourage les efforts et participe des replis identitaires. Venons-en brièvement au constat. La situation sociale étant partie polarisée dans les établissements publics à la rentrée 2021, la proportion d'élèves issus de milieux défavorisés est en moyenne de 37 4 % au collège. Mais si nous regardons en détails parmi ses élèves les plus défavorisés. On les retrouve pour 61% dans un dixième des collèges les plus défavorisés. Alors que les collèges les plus favorisés n'en accueille que 14,6%. En miroir, les 23,9% d'enfants issus de milieux très favorisés ne sont présents qu'à hauteur de 6,6% dans les collèges les plus défavorisés. Alors qu'ils sont près de 45% dans les 10% des collèges les plus favorisés. La différenciation sociale mesdames et messieurs les sénateurs, est encore plus marquée entre le public et le privé. La proportion moyenne des élèves de milieux défavorisés et de 42% dans le public mais seulement de 18% dans le privé et les écarts se creusent depuis le début des années 2000 l'IPS, l'indice de position sociale moyen dans le public hors éducation prioritaire et de 106 alors qu'il est de 121 dans le privé sous contrat. Ces constats implacables s'observe particulièrement au collège et il concerne à la fois l'enseignement privé sous contrat et l'enseignement public dans un contexte où l'écart entre les deux n'a cessé de s'accroître depuis plusieurs décennies. Afin de faire de l'égalité des chances et de la réussite de tous les élèves, une priorité. J'ai entamé un cycle de concertation et de consultation avec l'ensemble des acteurs concernés par le chant de la mixité sociale et scolaire. Les organisations syndicales représentatives de la communauté enseignante. De de l'enseignement public et privé sous contrat, les collectivités locales, les élus, les ministères partenaires joint un rôle essentiel les concertations avec les collectivités locales s'inscrivent dans le cadre de l'instance de dialogue entre le ministère et les collectivités locales que j'ai souhaité instaurer en septembre 2022 et je situe résolument ce cycle de consultations et de concertation dans une démarche Il nous faudra passer des bonnes intentions. À des solutions pragmatiques compréhensible et acceptable par tous. Pour cela, il n'existe pas, il est 7 évident de modèles clés en main les expériences menées, même les plus réussies n'ont pas vocation à être simplement mécaniquement dupliquer sans adaptation quel que soit le territoire ces ressources ou ses particularités. Il est de mon rôle de donner. Une impulsion de proposer des leviers d'action variées, ils existent et je ne doute pas que les acteurs seront sans dans Paris, voir en inventer d'autres. Le plus évident de ces leviers c'est bien évidemment la détermination de la sectorisation à travers la carte scolaire peut être d'ailleurs faut-il s'interroger avant. Avant cette étape sur le rôle joué par les politiques d'habitat et sur le choix géographique d'implantation des établissements scolaires. Le département de Haute Garonne que vous avez cité madame la sénatrice, qui a mené un travail résolu et réussi pour créer les conditions d'une mixité scolaire. Là par exemple pas hésité à détruire des établissements enclavé est connoté de longue date pour les reconstruire ailleurs. Si la prise en compte de l'objectif de mixité dans l'affectation des élèves des avec des secteurs multi-collèges est une solution qui porte ses fruits et qui moyennant explications famille. Prise en compte des temps de trajet ou des moyens de transport produit des effets assez vite mesurable. La fusion d'établissement voir la création de binômes de collège peu éloignés géographiquement avec des configurations variées ou des jumelages d'établissements permettent aussi d'améliorer l'hétérogénéité sociale des élèves, où nous avons repéré environ 200 binôme potentiels. L'implantation de d'offres de formation attractive dans les établissements défavorisés reste aussi un outil très efficace concernant les sections internationales par exemple on assiste en une année scolaire à une hausse de 3 à 8 points de l'IPS moyen dans les établissements où elles sont créées, 43 sections internationales nouvelles ont donc été créées dans des collèges d'éducation prioritaire en 2022, 16 autres le seront en 2023. L'absence de mixité existe aussi en milieu rural, il faut trouver des moyens particuliers d'action en rapprochant par exemple des établissements isolés de ce débours plus important par des projets communs ou des échanges pédagogiques. En parallèle, parce que la l'argent public finance aussi l'enseignement privé sous contrat, il est normal d'exiger de lui qu'il favorise aussi la mixité des élèves, en s'engageant dans une démarche contractualisé. C'est d'ailleurs ce que recommande le rapport du président Laurent Lafon et du sénateur Yves ou rendu en 2019 sur les nouveaux territoires d'éducation. J'ai donc entamer une discussion constructive avec l'enseignement catholique pour établir un protocole d'engagement qui j'espère sera signé dans quelques semaines, je mène aussi ce travail auprès des autres. Confessions disons ainsi qu'avec des établissements privés laïcs. Même si bien sûr il existe des a priori des préjugés, des volontés d'entre eux, soit représentations négatives et stigmatisons stigmatisante contre lesquels nous devons lutter et même s'il faut dire et redire que la mixité sociale ne fait pas baisser le niveau des élèves, il faut aussi entendre le soit des parents d'offrir le meilleur la seule réponse à cela, c'est aussi de renforcer l'attractivité des établissements publics pour permettre aux parents un choix rassurant. Je suis conscient et je ne nie pas les raisons qui poussent certaines familles à choisir soit de contourner la sectorisation soit de recourir à l'enseignement privé, parfois, pour certains au prix de sacrifices importants. Pardon je conclus en disant comme vous l'avez compris, faire de la mixité sociale, ce n'est pas remettre en cause la liberté scolaire ça n'est pas non plus faire gagner un camp contre un autre une catégorie contre une autre, c'est au contraire permettre l'enrichissement de tous ces permettre un socle commun pour tous, c'est assurer les conditions de l'altérité. C'est permettre de continuer à faire de la nation à faire de la France une nation je sais pouvoir compter mesdames et messieurs les sénateurs sur le soutien de tous ceux qui veulent faire vivre en actes la belle devise de notre République. Je vous remercie, le gouvernement aura la faculté s'il le juge nécessaire de répondre à une réplique pendant une minute l'oral. L'auteur de la question disposera alors à son tour du droit de répondre aux pendant une minute. Premier orateur, monsieur Pierre Jean Vergnes, Eulen pour le groupe les indépendants pour 2 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chacune et chacun d'entre nous a conscience de l'importance de faire vivre la mixité dans nos écoles de France. La mixité, elle permet de se confronter à la différence, quelle qu'en soit la forme. Elle permet d'apprendre à comprendre l'autre. Elle participe à former un citoyen. Mais le sujet de la mixité ne se pose pas pareil avec la même intensité selon les territoires. Chacun son expérience moi c'est celle d'un maire d'une commune rurale dans l'aine et j'imagine que l'enjeu et le sujet. N'est pas le même quand on est maire d'une ville centre ou des villes de banlieue. Et pourtant des décrochages des problèmes, des difficultés de mixité. Il y en a partout. Et évidemment il y a pas de classement à faire en la matière. Néanmoins. Les difficultés quand on est dans un territoire métropolitain grâce à la mobilité. Je veux dire au RER au métro au bus fait que vous avez accès à des lieux culturels. Enfin, pour faire simple le le le monde est devant vous et vous pouvez le voir. Or dans les territoires ruraux, soit vous êtes dans une famille qui a les moyens et l'organisation qui permet de se rendre dans ces endroits. Et des fois c'est la double peine. Vous avez les difficultés, vous êtes dans une famille où des fois il y a pas un permis de conduire. Vous êtes dans une famille où il y a pas les moyens de partir une journée où plusieurs jours pour se rend dans une capitale une grande ville pour s'ouvrir l'esprit cet éloignement ces difficultés ce manque de mixité n'est pas toujours pris en compte dans la mise en oeuvre des politiques scolaires et pour et pourrait pourtant faire la différence dans certains cas. Il s'agit de donner les mêmes conditions les mêmes chances. Les mêmes opportunités à chacun. C'est ça la vocation de l'école républicaine qu'sont en la matière, vos ambitions pour favoriser la mixité sociale dans les territoires ruraux et lutter contre les inégalités territoriales. Monsieur le Ministre. Merci, cher collègue, Merci monsieur le. Président me mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Vert de laine. Vous avez raison, la question de la mixité sociale ne se pose pas seulement dans les territoires urbains mais également dans les régions rurales cependant les problématiques. Scolaires dans les régions rurales sont un peu différentes des problématiques des territoires urbains. Globalement, les résultats scolaires dans les régions rurales avec des variations, il faut le reconnaître, sont des résultats corrects, voire même bon dans des départements très ruraux si je prends le cas de la Mayenne, par exemple les résultats scolaires en Mayenne. Sont de bons résultats scolaires. Néanmoins ce que l'on constate c'est plutôt une, un manque d'ambition ou en tout cas des difficultés à projeter ses résultats scolaires, dans des études post-bac qui impliquent éventuellement un un éloignement géographique de la région d'origine. Donc la question de l'éloignement à travers cet exemple est absolument centrale. En ce qui concerne les territoires ruraux. C'est pourquoi j'ai mentionné dans mon intervention la possibilité d'organiser des rapprochements entre établissements scolaires. Moyennement éloignées je dirais en tout cas éloignées de façon gérable par des modes de transport approprié j'ai. Également en tête. L'important, c'est l'intérêt des cordées de la réussite. Vous savez que 168.000 élèves sont aujourd'hui concernés. Nous visons un objectif de 200.000 élèves. Cordée depuis le supérieur au lycée

et. De la ville. Question qui va aussi impliquer. Les territoires ruraux et nous allons prendre notre temps pour aboutir à une refonte. En septembre. 2024. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je tiens d'abord à remercier mes collègues du groupe socialiste, pour l'inscription de ce débat essentiel à notre ordre du jour. Il y a beaucoup de choses à dire sur la mixité sociale et plus largement sur le sujet des inégalités à l'école. La France est l'un des pays de l'OCDE où l'origine sociale d'un élève pèse le plus sur son destin scolaire. Notre système éducatif et l'un de ceux qui reproduit le plus les inégalités, les inégalités sociales et ce depuis plus de 10 ans le manque de mixité sociale à l'école est un facteur aggravant des inégalités et sur ce point, la France est à la traîne, on assiste au développement d'une école à 2 vitesses, les établissements privés sont devenus l'un des moteurs de la ségrégation scolaire, en favorisant l'évitement de la carte scolaire pour les classes les plus favorisées. Selon une étude de la DEP à la rentrée 2021 40,1 % des collégiens du secteur privé sous contrat était issu des milieux scolaires très favori des milieux sociaux très favorisés contre 19,5% dans le public. Vous avez, Monsieur le Ministre, annoncé que la mixité sociale à l'école était l'une de vos priorités et nous nous en réjouissons tant votre prédécesseur a ignoré cette problématique dans ce cadre. Vous avez déclaré souhaité mettre en place un accord avec les établissements privés sous contrat et vous venez de le réaffirmer et il est vrai que le taux de boursiers dans l'enseignement privé sous contrat est actuellement inférieur à 10% et cela a à 10% et cela a été dit l'État et les collectivités territoriales subventionnent pourtant l'enseignement privé sous contrat à hauteur de 73%. Et donc la question des modalités de cet accord nous interroge quels en seront les termes, allez-vous enfin pondérer les subventions publiques au privé en fonction d'un ratio de mixité sociale acceptable en d'autres termes, allez-vous conditionner les aides aux établissements privés sous contrat à des taux de boursiers largement plus conséquents afin de cesser de financer sur données publiques la ségrégation sociale. Je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. que l'enseignement privé sous contrat. Sera impliqué dans cet effort de mixité tous les chercheurs qui ont travaillé sur cette question ont abouti à la même conclusion, si on ne n'implique pas l'enseignement privé sous contrat, les politiques de mixité sociale et scolaire. Ce seront sinon voué à l'échec. En tout cas très limités. Vous avez rappelé également que. L'État finance environ aux 3 quarts les établissements. Privés Privés sous contrat. Nous sommes donc en en négociation, en discussion avec le principal. La principale organisation qui regroupe l'essentiel des établissements privés je me réjouis de la, de la bonne volonté du secrétariat général de l'enseignement catholique ainsi que d'autres fédérations. Ou associations. Que j'ai pu consulter ces dernières. Semaines en effet, je crois qu'il y a 2. Écueils à éviter le 1er écueil consiste à finalement ne rien demander. Aux établissements privés sous contrat en échange de du financement dont nous parlons. Et laisser l'enseignement privé sous contrat libre d'agir comme il le souhaite. L'écueil inverse. Serait de faire passer l'enseignement privé sous contrat, sous les fourches caudines du public ce qui se heurterait à des difficultés très nombreuses à des résistances politiques très importantes. Il y a un espace. Entre ces 2 pôles si je puis dire, c'est l'espace de négociation par lequel effectivement nous avons des moyens d'agir, notamment. en modulant. Non pas la part fixe mais une part variable en quelque sorte, de notre subvention aux établissements publics privés sous contrat, mais c'est le cas aussi, j'insiste, des collectivités locales qui peuvent également moduler. C'est ce que le département de la Haute-Garonne et la ville de Paris ont

Monsieur le Ministre si la mixité sociale à l'école est si importante, c'est parce qu'elle un prérequis incontournable incompressible du vivre ensemble et le vivre ensemble ne se décrète pas. Il s'apprend il s'exerce en ce sens l'école publique est évidemment le lieu privilégié de cet apprentissage dès le plus jeune âge, l'école qui émancipe par le savoir et la culture bâti également un projet démocratique fondé sur des principes communs partagés et respectée par tous. Alors je fais partie de ceux qui pensent que l'école doit faire davantage pour la mixité sociale à ce titre, l'expérimentation des secteurs multi-collèges dans six établissements parisiens, dont les résultats sont positifs, va dans le bon sens mais la mixité sociale à l'école n'est pas le seul fait de l'école, vous le savez, la carte scolaire des écoles maternelles et élémentaires et déterminé par les conseils municipaux et celle des collèges par les conseils départementaux par ailleurs nos écoles sont des réalités physiques des réalités urbaines. Elle s'insère dans un environnement urbain qui agit lui aussi sur la mixité sociale. Les politiques de l'urbanisme et de l'habitat ont donc également un rôle à jouer. quel rôle votre ministère pourrait-il avoir dans la nécessaire coordination entre les différents acteurs qui de près ou de loin agissent sur la mixité sociale à l'école.

le travail de l'éducation nationale et d'autres ministères. Je pense en particulier à celui de la ville et du logement et nous sommes en en au travail avec mon collègue Olivier Klein dans la perspective que j'indiquais précédemment, c'est-à-dire celle de la refonte en tout cas de retouche et d'un travail sur la carte de l'éducation prioritaire. Cette carte est en effet fondée sur des données qui remontent à 2011, la carte elle-même datant de 2015, or les changements sociologiques. urbain de la société française impose certainement de retoucher de repenser cette carte en particulier pour les établissements de REP. Les établissements href plus sont d'une certaine façon très immobile, puisqu'ils sont inscrits dans des quartiers défavorisés qui malheureusement n'ont pas changé de façon importante depuis 10 ans. En revanche, les quartiers REP. Un peu plus intermédiaires. Ont subi ou ont connu des des changements sociaux important avec par exemple à Paris des phénomènes de de gentrification qui ont profondément modifié ses quartiers et puis il y a aussi des des régions ou des, ou des secteurs qui ont été un peu oubliée. En 2015, bref il faut repenser cela en cela en lien effectivement avec. Les quartiers prioritaires de la ville. Sur lesquelles travaille le ministère de la ville et du logement. J'ajoute enfin un point très important c'est le fait que. En dépit des pesanteurs qui sont des pesanteurs urbaine et sociale, nous pouvons néanmoins prendre des initiatives. Pour aller au-delà des frontières sociales, je pense en particulier à ce qui a été fait à Toulouse puisqu'on déplace les élèves des collèges du quartier du Mirail vers des quartiers centraux et donc en dépit de la pesanteur sociologique du quartier du Mirail. On peut obtenir des résultats scolaires indépendamment en quelque sorte d'un bâti urbain et de données sociologiques existantes. Merci, monsieur le Ministre. Pas de réplique. La parole est à monsieur Yan Chantrel. Pour le groupe socialiste. Pour 2 minutes. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Comme ça a été rappelé par par différents intervenants intervenantes notre dans notre pays, l'enseignement privé sous contrat est subventionné par l'État et les collectivités territoriales à hauteur de 73%. C'est près de 10 milliards d'euros qui chaque année sortent des caisses publiques pour financer le privé alors que le public souffrent d'un manque de moyens. Chronique le privé continue de profiter de, de nouveaux effets d'aubaine, comme avec la loi Carle en 2009 et la loi blanquette en 2019. Or, cas unique au monde. Ce financement public du privé se fait pratiquement sans aucune contrepartie. Ces établissements échappe à la carte scolaire et leur recrutement reste opaque, on ne sait pas quels critères sont retenus pour sélectionner les élèves. Tout le monde finance le privé mais tout le monde n'y a pas accès car le privé pratique l'exclusion sociale de fait en juillet 2022, vos services soulignait que l'écart entre la proportion d'élèves très favorisés dans le privé et le public s'était creusé de près de 10 points en 20 ans. La publication des IPS en janvier a confirmé l'embourgeoisement de plus en plus marquée du privé à Paris. De chercheur Julien Grenet et Youssef Souidi ont montré que le privé ne compte que 3% d'élèves défavorisés, contre 24% dans le public il est là le véritable séparatisme contre lequel nous devons lutter avec acharnement. Pire, une étude de 2014, mené par Loïck du parquet Thomas Dati et Pascal Petit au moyen d'une expérience. Inspirer de la méthode du testing a démontrer qu'il existe à l'entrée des établissements scolaires privés une sélection ethnique en tant que chercheur, vous serez vous aussi sensible que moi la pertinence de ces travaux. Ce constat. Je sais que vous le partagez vos convictions, nous les connaissons. Monsieur le Ministre, nous sommes prêts à vous soutenir contre tous les conservatismes. Si vous prenez des mesures à la hauteur de l'urgence. Mais êtes-vous prêt Monsieur le Ministre à introduire au niveau national, un système de bonus malus similaire à celui mis en place par le département de Haute-Garonne. Parce que vous n'avez pas été précis suffisamment précis sur ce point pour moduler les crédits pédagogiques versés aux établissements en fonction de leur niveau de mixité sociale en fait ça reviendrait à prendre l'argent au leur faire que privé qui ne jouent pas le le jeu de la mixité sociale, pour le donner au public. Merci monsieur Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Chantrel. La question du financement du privé. En tout cas du privé sous contrat que vous abordez. Je souhaite le faire par la concertation et je souhaite le aboutir à un protocole d'accord avec des objectifs précis non pas un protocole vague mais avec des objectifs précis et je note la bonne disposition de nos interlocuteurs. Du privé sous contrat parce que. Les temps ont changé aussi la publication des IPS à jouer aussi son rôle et nous avons quelques moyens de pression, si je puis dire. J'ai mentionné la question des collectivités. Locales qui peuvent en effet agir, c'est le cas du département de Haute-Garonne. C'est le cas aussi de la ville de Paris nous même nous pouvons agir Les moyens. D'enseignement. L'allocation de poste lorsque des demandes sont faites par le privé sous contrat peut aussi être un facteur. De pression si je puis dire sur les établissements de manière à ce que il s'engage dans des politiques résolu. De mixité sociale et Je dis, mixité sociale et scolaire parce que. Un simple objectif de fixation d'un pourcentage de boursiers certes intéressant ne doit pas aboutir à ce que les établissements privés sous contrat aille chercher dans le public, les meilleurs élèves. Boursiers en quelque sorte en privant les établissements publics de leur têtes de classe. Il faut donc veiller à une mixité scolaire qui ajoute au facteurs purement social, d'autres facteurs, par exemple. Les élèves en situation de handicap puisque le taux d'élèves en situation de handicap et plus. Significativement plus bas dans l'enseignement privé sous contrat également des élèves dont les résultats scolaires soient répartis je dirais sur l'ensemble du spectre. C'est donc à tout ce travail que nous sommes attelés pour aboutir à un protocole aux alentours du 20 mars. Merci monsieur le ministre madame Céline ne brûle hein pour le groupe CRCE pour 2 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cela a été dit l'école française est l'une des plus inégalitaires des pays de l'OCDE, il y a donc besoin de mesures structurelles et pas seulement de ce que je qualifierais de cosmétiques. Prenons l'exemple du lycée Claude Monet au Havre depuis 2018. Celui-ci a perdu l'équivalent de 8 postes alors qu'il a accueilli 35 élèves de plus sur la période l'indice de position sociale de cet établissement à baisser d'année en année atteignant actuellement 92. 9. Alors que le lycée privé Saint-Joseph située à 150 mètres à lui un IPS de quasiment 138 face à la dégradation de la situation sociale des élèves de l'établissement public. Il va falloir davantage couvrir des formations attractive ou inciter les parents d'élèves du lycée privé à inscrire les leurs enfants à Claude Monet. Monsieur le Ministre de la communauté éducative vous demande non pas un énième artifices mais des moyens pour pallier les conséquences des inégalités socio-économiques que subissent certains élèves au travers d'un renforcement de l'action pédagogique et éducative. Ça n'a pas tout à fait ce que vous faites dans les attributions de dotation horaire globale actuellement examiné dans le secondaire, ni dans les mesures de carte scolaire en primaire puisqu'en REP et en REP plus ou dans le rural isolé. Où il existe aussi de nombreuses difficultés sociales, nous continuons à perdre des moyens d'enseignement. Allez-vous mieux tenir compte de la réalité sociale dans l'allocation des postes qui s'apparente aujourd'hui trop souvent à une gestion comptable. Merci. Merci, monsieur le Ministre. Merci monsieur le président. Merci madame la sénatrice. Brûle hein. Je ne connais pas la. Situation spécifique du lycée Claude Monet du Havre mais je, je la regarderai. Et. Croyez bien que. Les réponses que vous. Attendez, ne relève pas simplement. De. Formation attractive il y a tout un éventail toute une palette. Y compris la question de la sectorisation que j'évoquais précédemment, qui ne concerne pas l'an l'établissement privé auquel vous faites allusion, mais qui peut concerner un et un autre établissement public. Dans le voisinage ou en tout cas dans la ville du Havre. La question en fait.

publics défavorisés a gardé des élèves qui sinon. Vont ailleurs, et en particulier dans l'enseignement privé sous contrat dans le lycée auquel vous faites allusion. Il est donc intéressant, utile de réfléchir à la meilleure manière de conserver ses élèves et des expériences très intéressantes, ont été menées un peu partout en France, qui indique bien que des formations d'excellence peuvent donner de bons résultats, ça peut être une classe de type préparation. Aux études supérieures de type Sciences Po par exemple par un conventionnement avec un institut d'études politiques, ça peut être une section internationale comme je l'ai mentionné quant aux moyens d'enseignement ils sont directement dépendants de des effectifs scolaires et nous veillons à ce que le taux d'encadrement en dépit de la baisse des moyens d'enseignement dans certaines régions s'améliore et ce sera le cas dans le département de Seine-Maritime. Merci. Une réplique. Merci monsieur le président. Vous venez d'indiquer Monsieur le ministre, et c'était le sens même de ma question, que l'allocation des moyens et quasiment exclusivement liées aux effectifs. ce cours sur quoi je voulais vous interpeller, c'est comment peut-on prendre en compte la situation sociale des établissements pour renforcer les moyens d'éducation. Par ailleurs, je trouve que dans la palette des propositions que vous faites vous mettez beaucoup à contribution les collectivités pour assurer la mixité sociale. Nous connaissons tous, ici, dans quelle situation. Elles sont aujourd'hui. Et enfin je suis inquiète sur ce qui pourrait s'apparenter dans ce que vous avez proposé aussi à d'éventuels regroupements d'écoles dans les centre-bourgs alors que l'existence d'une école rurale avec un maillage très fin du territoire est aussi un gage de rire. Monsieur le président, madame la sénatrice brûle hein. Les moyens d'enseignement ne dépendent pas que des effectifs, ils dépendent aussi de l'IPS de l'indice de positionnement social, ils dépendent aussi de l'éloignement. Et on calcule et donc il y a des variations qui peuvent être complètement indépendante des effectifs. Stricto sensu, et c'est un travail que les directions académique mène chaque année en collaboration d'ailleurs et en échange avec les. Élus. Sur. Le point que vous. Mentionnez. Il ne in fine et là je j'attire simplement votre attention sur l'intérêt du maillage mais aussi sur le fait que. Dans le secondaire, tout au moins les bombes, les meilleurs résultats scolaires ne sont pas enregistrées par les tout petits établissements il y a pas de lien entre la taille des établissements et la réussite scolaire ou plutôt la petite taille des établissements et parfois. N'est n'est pas là la la meilleure recette ou en tout cas la garantie. De résultats scolaires convenable. On a il y a une taille critique a pensé pour les établissements qui est important pour la réussite de nos élèves. Merci. Oui alors J'entends que vous prenez en compte. Monsieur le Ministre. Les IPS dans la location de moyens et donc nous allons argumenter sur un certain nombre de situations qui vont j'espère permettre qu'on attribue davantage de postes et de des HUG aux aux établissements en question et j'insiste vraiment sur le maillage scolaire en milieu rural qui favorise la réussite des élèves, notamment parce que dans les communes rurales autour de l'école se nouent des relations sociales des associations un vivier qui contribue aussi à la réussite et ça me semble très important. la parole est à monsieur Claude Kern pour le groupe Union centriste pour 2 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors que le postulat de départ est clair, le premier article du code de l'éducation, vous l'avez rappelé rend la mixité obligatoire dans l'enseignement primaire et secondaire. Près de 50 ans plus tard, force est de constater que cet objectif est loin d'être atteint et reste malheureusement un véritable sujet, le rapport de la Cour des comptes de décembre 2021, constate d'ailleurs que la possibilité pour chaque enfant d'accéder, quelles que soient ses origines, aux mêmes conditions de scolarisation n'est pas garantie. C'est un frein à l'efficacité générale de l'école qui reste segmentée et dont l'impact négatif en termes d'accès au savoir, à la culture et tout simplement d'appartenance à une même nation. Alors la question, la simple quel plan comptez-vous mettre en oeuvre aujourd'hui pour rendre concret. L'objectif de mixité sociale fixées dans le code de l'éducation. Par ailleurs et concernant l'enseignement privé sous contrat, vous avez récemment les efforts à envisager alors afin qu'ils participent à une plus grande mixité sociale. Ah quels efforts pensez-vous et concrètement, quelles sont vos leviers de mise en Oeuvres, sachant que la loi reconnaît à ces établissements à caractère propre enfin quel bilan et enseignement tirez-vous des réformes mises en place que ce soit pour rendre l'école plus juste, avec la loi de refondation de l'école mais également concernant la sectorisation dans le secondaire Somme, l'assouplissement de 2007 n'a in fine est pas modifier la composition sociale des collèges à l'échelle nationale vouloir évaluer l'efficacité et corriger le cas et chez le cas échéant les faiblesses d'une politique publique en proposant des alternatives demande du courage politique. Un message clair et fort massivement compris et soutenu non l'impulsion ne peut venir que de l'État de manière transversale qu'sont à la matière vos objectifs et la manière dont vous amorcerait le changement nécessaire pour permettre à l'enseignement obligatoire de jouer pleinement son rôle intégrateur. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. un seul levier mais une palette. De levier qui peuvent être appliquées selon avec des variations selon les territoires. Il les réalités locales. C'est pourquoi la méthode consiste à proposer une palette. que les recteurs et les lectrices en lien avec les collectivités seront en charge d'utiliser souplement voire d'en inventer d'autres. Afin d'obtenir des objectifs que nous leur fixeront avec une progressivité annuel. Parmi ces leviers, j'ai mentionné la question de l'enseignement privé sous contrat en effet et j'ai indiqué que nous sommes dans une démarche de négociation pour obtenir un protocole. Nous avons des moyens d'action en effet j'ai mentionné la question des postes, j'ai mentionné aussi la question des bonus malus en quelque sorte, que les collectivités peuvent appliquer nous-mêmes aussi. Via le poste 139, avons des moyens. D'action en matière d'allocations de fonds au-delà de ce que nous devons bien entendu à l'enseignement privé sous contrat qui assure une mission de service public. La question de la sectorisation. C'est une question qui a fait l'objet de beaucoup de travaux et beaucoup de, de réflexion, en effet depuis. Plus de de 15 ans. Je vous invite à regarder ce qui a été fait récemment à Paris Dans le cadre d'Affelnet. Pour l'affectation des lycéens pour l'entrée en en seconde et qui a donné des résultats tout à fait probant avec des établissements qui recevait peu d'élèves boursiers qui en reçoivent. Désormais Désormais beaucoup plus, c'est le cas de certains s'établissement très prestigieux et à l'inverse, des établissements qui avait un très fort taux de boursiers dont la population scolaire est désormais plus équilibré avec l'aide des chercheurs avec les travaux et les statistiques de la Nous avançons et nous avons une connaissance beaucoup plus fine. De la carte scolaire, qu'il y a une quinzaine d'années. La principale injustice de notre pays, c'est le déterminisme familial, la trop faible mobilité sociale. La réponse se trouve dans l'école. L'orientation ces mots, c'est Emmanuel Macron qui les a prononcés pour ses voeux aux Français en 2023. Le secteur privé compte 40% d'élèves très aisés, contre 20% dans le public, 42% des élèves du public sont issus de milieux sociaux défavorisés. Ils ne sont que 18% dans le privé. ces écarts ne font que se creuser à un rythme accéléré depuis les années 2010. Vous avez dit vouloir impliquer l'enseignement privé sous contrat, dans la poursuite de l'objectif de mixité sociale consubstantielle à celui d'égalité des chances. Le taux de boursiers dans les écoles privées sous contrat est actuellement inférieur à 10%. Trop faible au regard de la composition sociale de nos effectifs colère selon vos propres mots. L'intégration, vous venez de le rappeler, depuis la rentrée 2022 des lycées Louis-le-Grand et Henri-IV. Dans le système d'affectation a fait le Net 100 prometteur leur candidat parisien ne sont plus recrutés sur dossier mais en fonction de leur proximité géographique et des caractéristiques sociales des quotas d'élèves boursiers sont désormais appliquées et parmi les secondes. La part des élèves de catégories moyennes et défavorisés est passé de 13 à 29% à Louis Legrand et de 12 à 22% à Henri IV. L'entrée des deux lycées dans a fait le Net semble avoir eu un effet incitatif sur les candidats puisque maintenant % sont plus nombreux à avoir candidaté par rapport à l'an dernier et issus de collèges plus divers. Alors. Jacques Attali, devant notre délégation à la prospective a recommandé entre 20 et 30% d'élèves issus de familles défavorisées dans tout l'établissement Êtes-vous prêt à imposer un niveau de mixité sociale équivalents dans tous les établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés sous contrat et comment. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur. Fier, vous avez en effet. Souligné l'écart qu'il y a entre un taux de boursiers inférieur à 10% dans la saignements privé sous contrat et un taux de boursiers avoisinant 29%. Dans l'enseignement public c'est globalement un rapport de un à 3, c'est un écart qu'il faut réduire d'où le protocole que j'espère nous allons pouvoir signer dans quelques semaines avec des engagements précis de la part des établissements privés sous contrat et je réitère la tension et et l'intérêt de. Leurs organisations représentatives. Pour ces questions, nous avons un certain nombre de points à à régler et il y a la question notamment de la restauration scolaire, qui pose un certain nombre de de de problèmes mais nous pouvons avancer, y compris avec l'aide des collectivités, vous avez mentionné le cas des lycées Louis-le-Grand et Henri IV très justement je souligne dans la réforme d'Affelnet que des lycéens de Louis-le-Grand par exemple peuvent venir de quartier assez éloigné du lycée Louis-le-Grand et pour cause, parce que le quartier du lycée le plus grand ne garantit pas une mixité sociale. Tous très très intense et donc on utilise les moyens de transport. Très dense à Paris en particulier la ligne du RER B pour acheminer vers le lycée Louis-le-Grand des. Élèves qui sont géographiquement relativement éloigné qui habitent par exemple dans le nord de Paris mais qui peuvent se rendre au lycée Louis-le-Grand en une demi-heure environ et donc c'est moins la proximité géographique qui compte que le temps de transport ce qui. Offrent beaucoup de possibilités dans une ville comme Paris, compte tenu de la densité de ces moyens de transport donc. La la réforme d'Affelnet a donné d'excellents résultats. Ça nécessite un travail extrêmement faim puisqu'il faut faire des calculs de mode de transport et donc la carte peut prendre une allure assez baroque, si je puis dire, mais c'est à cette condition qu'on a pu obtenir des résultats tout à fait probant pour des lycées qui était en quelque sorte hors normes par le recrutement mais aussi par le résultat scolaire. Et Monsieur le Ministre, la parole est à monsieur Max Brisson pour le les républicains pour 2 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre voudrais d'abord rappeler une réalité. La France enregistre de bien mauvais résultats concernant la réussite scolaire de tous ses élèves certes particulièrement ceux issus des milieux défavorisés mais aussi les autres. Dans ton soutient donc toute initiative visant à assurer la performance scolaire et l'égalité des chances. Il ressort de vos premières annonces que vous souhaitez principalement revoir la sectorisation et ouvrir davantage en ce moment privés à la mixité sociale, pourquoi pas. Mais le risque sera grand de renforcer l'incompréhension des parents, des parents et la mise en place de stratégies d'évitement, sans apporter de réponse globale et durable à la question de la réussite de tous les élèves. En réalité, nous ne poursuivrons pas le même objectif vous parler de mixité sociale. Nous parlons d'égalité des chances et de réussite scolaire. Pour y parvenir. Ne faudrait-il pas mieux nommé dans l'établissement. Ah besoins éducatifs particuliers des enseignants expérimentés l'affectation quasi exclusive de professeurs fraîchement issues des Inspé ou même de formation accélérée de 48h heures.

pour laisser aux acteurs de terrain, des marges de manoeuvre nécessaires et les moyens d'assurer l'égalité des chances, ne faut-il pas en fait instaurer un véritable service public du soutien scolaire. Épaulé par la création d'une réserve éducative. Voilà les propositions que je souhaitais formulé et dont nous reparlerons. Qu'en pensez-vous monsieur le ministre. Merci monsieur le ministre. réussite de tous les élèves d'ailleurs des études il était fait allusion aux travaux de Monsieur Grenet. Précédemment montre que. Les établissements où il y a de la mixité, où l'on crée de la mixité. Donc par exemple à Paris ou à Toulouse puisqu'on a cité c'est de ces deux villes sont des établissements où les élèves défavorisés. Voient leurs résultats progresser d'ailleurs pas dans des proportions spectaculaires. Il n'y a pas de baguette magique. En la matière, tandis que les élèves favorisés ne voit pas du tout leur résultats baisser, donc ça ne se joue pas au détriment des uns par rapport aux autres ce que les travaux montrent c'est 2 choses, d'une part que les élèves défavorisés voient leur ambition scolaire et post-bac décuplée. Ils ont des perspectives, il il il se projette d'une manière très différente de. Leur situation précédente, d'autre part les réseaux. Sociaux les réseaux d'amitié entre les élèves se reconfigure. Autrement dit les élèves ce mélange entre eux ils ne forment pas des groupes qui seraient des groupes séparés et qui obéirait aux logiques. Scolaire Scolaire précédente mais on a des reconfigurations sociales tout à fait intéressante et donc il faut penser la mixité comme un facteur de réussite et pas comme quelque chose qui viendrait en quelque sorte embarrassé cette réussite sociale. Je vous rejoins et nous aurons l'occasion de reparler sur la question de la formation des enseignants. Nous avons besoin d'enseignants mieux formés, puisque la France est un pays où la formation académique et longue importante plus long qu'ailleurs, mais la formation au métier et courte, ce qui est paradoxal, compte tenu du fait que l'on envoie ensuite les enseignants dans des écoles ou des établissements où on réclame où on attend une formation importante au métier, nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci Monsieur Bresson. Oui, Monsieur le Ministre, je ne crois pas que c'est en permettant quelques élèves de milieux défavorisés de se retrouver à Pierre de Fermat, où a lieu le grand qu'on réglera le problème de la mixité sociale et des difficultés des élèves issus des milieux défavorisés, je le répète, ce n'est pas en tentant d'imposer la mixité sociale à tout prix par la sectorisation rigide et les quotas que nous pourrons faire progresser le niveau scolaire des élèves les plus éloignés de la réussite, nous le ferons par la différenciation de politique éducative sur le terrain dans ces établissements qui passe par une nouvelle approche contractualisé des ressources humaines et de l'affectation des moyens dans nos territoires. Merci, monsieur le Ministre. Monsieur le sénateur Brisson. Il n'y a pas de, je ne vois pas de contradiction là non plus il ne s'agit pas de quelques élèves qui. Viendraient simplement masqué le reste à Toulouse par exemple en ce qui concerne le quartier du Mirail, ce sont plusieurs centaines d'élèves qui ont été envoyées dans 7. Collèges principalement de centre-ville mais aussi. De bordure de Toulouse on a donc un nombre. Très important de ses élèves qui ne sont pas que les meilleurs élèves des quartiers du Mirail, mais avec une mixité scolaire importante. Donc c'est une expérience qui mérite d'être regardé de près. Par ailleurs, il y a, j'insiste sur ce point l'importance d'implanter et de et de valoriser des établissements défavorisés avec des filières d'excellence avec aussi des travaux sur le bâti scolaire, pour revaloriser des établissements qui sont en effet problématiques ou délaissés. Merci ce Bresson. Et alors, Monsieur le Ministre, je ne vous embêterai pas davantage que caractère cosmétique de ce dont vous parlez. Par contre je vous repose la question, est-ce qu'on on nous en reparlerons. Est-ce, quand est-ce que nous arrêterons. De nommer dans d'affecter dans les établissements des quartiers les plus difficiles, où la population a des besoins éducatifs particuliers les professeurs les plus jeunes, les moins expérimentés. Ce qui sort des Inspé, les vacataires qui sortent de quelques heures de formation, quand est-ce qu'on n'a pas, on va réfléchir à une nouvelle politique des ressources humaines, amenant dans ces établissements, des professeurs chevronnés expérimenté et capable justement de sortir le plus grand nombre des difficultés scolaires, dans lequel il se trouve. Merci, cher collègue, la parole à Marie-Pierre Monnier. Pour le groupe socialiste pour 2 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la question de la mixité scolaire se pose différemment en agglomération et dans les territoires ruraux où les établissements scolaires sont plus éloignés les uns des autres, limitant ainsi l'impact de la ségrégation résidentielle les stratégies d'évitement des familles, la mixité est une réalité bien plus tangibles dans les écoles, collèges et lycées de nos communes rurales où le vivre-ensemble existe de fait une raison supplémentaire de leur accorder les moyens de fonctionner dans des conditions correctes et de maintenir leur ancrage territorial. Car sur le terrain on observe une montée en puissance des écoles privées rurales notamment hors contrat qui pourrait remettre en cause ce fragile équilibre. Or, nous payons aujourd'hui très chère. Les suppressions de postes acté lors du vote du budget 2023 notamment dans le 1er degré dans la Drôme. Plus de 40 fermetures de classe vont avoir lieu essentiellement dans les communes rurales. Victime d'une logique comptable. Que prévoyez-vous pour maintenir des conditions d'enseignement à la hauteur dans ces territoires, la situation des lycées ruraux doit également appeler votre attention car la mise en oeuvre de la réforme du lycée a mis à mal leur attractivité. Nous l'avions pointé dans notre rapport de bilan des mesures éducatives du quinquennat. Avec mes collègues Annick Billon et Max Brisson. Les lycées ruraux se trouve en raison de leur dotation globale horaire limité, contraint de faire des choix entre spécialités et options proposées. Cela incite des élèves au départ de leur établissement. Le gouvernement a-t-il prévu de renforcer les moyens qui leur sont consacrés. Afin de garantir une offre éducative homogène une égalité d'accès aux renseignements facteur clé de la mixité sociale. Merci, monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice. Mounier. La question. Du du rural, à mon sens, ne peut pas et au sens des données dont nous disposons, ne peut pas être abordé en laissant entendre que les écoles rurales seraient sous-dotée par rapport aux écoles urbaines, c'est même le contraire en réalité avec un taux d'encadrement qui est souvent meilleure dans les écoles rurales. Sont dans les établissements ruraux et cela concerne 35% des écoles. Il est vrai que il y a une baisse des moyens d'enseignement. Pour la rentrée 2023 qui correspond malheureusement si je puis dire. À une baisse des effectifs scolaires. Mais la baisse des moyens d'enseignement n'est pas fait arithmétiquement ou en proportion de la baisse des effectifs scolaires de telle manière à ce que le taux d'encadrement s'améliore. Par ailleurs, nous regardons les situations délicates au cas par cas puisque d'ici au mois de juin nous allons procéder à un certain nombre d'ajustements dans les différentes académies. En ce qui concerne les lycées, la réforme des lycées n'a pas restreint le choix

Numérique sciences informatiques et des sciences de l'ingénieur puisque nous souhaitons accroître le nombre d'élèves qui se dirige vers les voies technologiques mais je souligne la variété des offres et qui est et et le fait que. L'existence de ces cette cette spécialité au moins permet tout de même un choix très large plus large en réalité que la situation précédente. Monsieur le Ministre, Madame. Moi Moi je voudrais revenir sur les sommes puissions de postes parce qu'on a bien le sentiment que c'est vraiment proportionnellement au nombre d'élèves que ces faits moyenne de de d'élèves par classe primaire ses 21,9 en France, en Europe, c'est 19 IV et dans nos classes rurales après fermeture au monde souvent 24 25 26. Ça c'est quand même quelque chose qui rend l'égalité Vous avez dit tout à l'heure que les directions académique négocie avec les élus, mais le font avec ce qu'on a voté au PLF c'est-à-dire avec pas grand chose en gros à Grenoble c'est 0 postes et la Drôme a dû rendre 11 postes et vous avez parlé de trajet raisonnables, ça, ça m'interpelle beaucoup de regroupements. On n'a pas envie de voir revenir le 6 squatter et je vous rappelle

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je souhaite d'abord remercier Sylvie Robert et son groupe politique à l'initiative de ce débat un débat sur l'école. Alors je pense aussi ce soir à la famille aux collègues et aux élèves d'Agnès Lassalle sauvagement assassinée dans son établissement scolaire. Monsieur le Ministre, 43 nouvelles sections internationales devait être ouverte à la rentrée 2022 dans les collèges les plus défavorisés. Ce dispositif bilingue qui propose d'accueillir des élèves français et étrangers dans une même section est un des deviez pour actionner favoriser améliorer la mixité sociale à l'école. Il permet aux élèves de bénéficier d'un total de 6h de cours supplémentaires par semaine, 2h d'histoire-géographie ou de mathématiques dans la langue de la section 4h de lettres étrangères. Monsieur le Ministre, mercredi dernier, vous avez affirmé votre volonté de multiplier les ouvertures de sections internationales dans les collèges et lycées défavorisés pour assurer ses 6h de cours hebdomadaires, les professeurs en poste devront être mobilisés et de nouveaux professeurs devront être embauché dans certaines académies. Or, les enseignants n'ont jamais été aussi nombreux à quitter leurs fonctions en 2008, il représentait 0,05% des effectifs aujourd'hui près de 3. cela vient s'ajouter aux démissions survenant après quelques semaines ou quelques mois d'exercice de certains certains enseignants contractuels recrutés à la rentrée 2022 pour pallier aux 4000 postes vacants de professeurs titulaires. Face aux difficultés de recrutement et à la crise d'attractivité du métier, comment entendez-vous, Monsieur le Ministre, garantir l'effectivité de ces sections internationales. Je vous remercie. Merci monsieur le président. Merci madame la sénatrice Lyon en effet la l'ouverture de sections internationales. Donnent de, de bons résultats. Je l'ai mentionné avec la hausse d'une année sur l'autre. De l'indice de positionnement social, ce qui est évidemment très bon signe pour des établissements défavorisés. C'est pour cela que nous n'ouvrirons des. Sections internationales que dans des établissements défavorisés pour rattraper en quelque sorte. Un retard y avoir des effets. Importants. En matière de moyens, il faut considérer que l'ouverture d'une section internationale commence par la classe de 6ème et puis ensuite progresse 5ème 4ème 3ème et donc la répartition des moyens ne se fait pas. dans le cadre du collège sur l'ensemble immédiatement sur l'ensemble des quatres années mais. Est en quelque sorte réparti d'une année à l'autre, ce qui permet. D'envisager l'ouverture de ces sections internationales de façon. Correcte, Correcte, j'allais dire, en dépit des difficultés, vous avez raison de le faire. Des difficultés de recrutement que nous avons dans le secondaire. Ces difficultés de recrutement sont inégales selon les disciplines. Elles sont fortes du côté des lettres modernes par exemple du côté de l'allemand aussi. Moindres mais tout de même du côté des mathématiques, de la physique chimie ou de la technologie mais nous avons choisi de faire un effort particulier dans ces établissements défavorisés et donc. D'y consacrer les moyens nécessaires à la rentrée 2023, nous ouvrirons 16 sections internationales supplémentaires et nos calculs. Démontrent que cela est possible. J'aimerais faire plus mais cela est possible avec 16 sections internationales supplémentaires. Le taux de démissions auquel vous faites allusion. Pour les enseignants. Contractuels et tu. En effet, une préoccupation et c'est pour cela que nous avons un programme sur le long terme, de formation des enseignants contractuels 87% des enseignants contractuels à la rentrée 2022 avait déjà enseigné l'année scolaire précédents. Ils n'ont pas été engagé ou embaucher embaucher à la dernière minute. En tout cas dans leur grande majorité, nous avons beaucoup d'enseignants contractuels qui ont une expérience parfois importantes sur plusieurs années. Merci réplique. Il y a 10 secondes. Merci, monsieur le Président bon écoutez. Vous parler de moyens vous parlez. Monsieur le ministre, en disant qu'il y a peu de risque de précarisation, je n'en suis pas convaincu. Vous allez mettre les moyens. Ce serait intéressant quand même d'avoir. Un retour sur ses investissements qui pourraient être mis et qu'on voit l'efficacité des deux par rapport. Aux objectifs fixés. Je je je reste sceptique à ce stade. Merci Monsieur Olivier Paccaud pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre. Il n'y a ni mauvaises homme ni mauvaises herbes, il n'y a que de mauvais cultivateur, écrivait Victor Hugo, avant que Jules Ferry n'édifie l'école républicaine comprenant que pour moissonner le bonheur public, il faut d'abord en semer les germes dans la jeunesse en rendant l'école laïque, gratuite et obligatoire pour tous la 3ème République poursuivait l'ambition de façonner des citoyens libres instruisez éclairé unis par des valeurs partagées dans le grand creuset social scolaire pendant des décennies, la République a fait de l'école, sa Pierre angulaire y plaçant toute son essence alors même que les divisions qui traversait la France était peut être plus vive qu'aujourd'hui l'école a donné une instruction solide à tous distinguer les plus méritants et offert à une république jeune hésitante un corps social cohérent et soudé derrière elle l'école alors cimenter la nation. Aujourd'hui elle si lézardes preuve de ce malaise, l'enseignement privé, donc on a beaucoup parlé ne sait jamais si bien porté et certainement pas pour des raisons religieuses. Ce que recherchent les parents d'élèves dans le privé d'aujourd'hui. C'est l'école publique d'hier. Ou le travail, la discipline, l'autorité du maître étaient les points cardinaux. Comment s'en étonner quand le niveau de ses élèves s'effondre. Quant au temps des hussards noirs a succédé celui des contractuels recrutés en job dating. Quand la carte de l'éducation prioritaire oublie les 3 quarts du pays. L'enjeu de la mixité sociale à l'école est capital pour empêcher l'avènement d'une société archipel mosaïque de groupes antagonistes, refusant de faire nation ensemble la non mixité sociale couve les séparatismes de demain la mixité elle forge le sentiment d'appartenance à une communauté de destin Lyon de toute société. Monsieur le Ministre, la première Pierre d'une vraie mixité sociale n'est-elle pas le retour à certains fondamentaux pédagogique, le travail, la discipline, le respect de l'enseignant. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur Paco. Je ne serai pas celui qui mettrait de côté ou qui d'évaluerait l'importance de l'effort, du travail et du mérite. Bien entendu et. De ce point de vue là, j'ai réintroduit par exemple les mathématiques en classe de première, dans la filière générale. Ça réclame des efforts supplémentaires, y compris pour les élèves qui n'ont pas ou peu d'appétence pour les mathématiques, pour ne prendre que cet exemple nous sommes attelés à faire du cours moyen et de la sixième un moment essentiel quant à revenir ou quant à voix quant à avoir pour l'école de jadis, permettez-moi en tant qu'historien d'être un peu sceptique. Car en effet si l'école de jadis, peut avoir un charme particulier en 2023. N'oublions pas que pour l'immense majorité des enfants ce qui étaient issus des couches populaires, l'école, ça reste s'arrêtait au certificat d'études, très peu étaient les élèves qui poursuivait au lycée. Jusqu'en, jusqu'au Baccalauréat vers 1960. Le pourcentage d'élèves ayant le bac était de 10%. Je ne regrette pas particulièrement ce temps là donc le le la trajectoire historique du XXe siècle, ça a été celle de la massification de l'école, c'est-à-dire de l'entrée. Je suis sûr que vous êtes en accord avec cela. De l'entrée au collège et de l'accès au lycée et puis ensuite notre enjeu aujourd'hui ça n'est plus celui de la massification c'est celui de la démocratisation, on peut dire, c'est-à-dire de faire de telle sorte que. Les élèves et un accès égal méritocratique à toutes les filières, que ce soit d'ailleurs des filières d'excellence dans le monde professionnel ou que ce soit des filières d'excellence dans les universités et plus tard dans. La vie professionnelle. Cette question là elle est allée centrale. Et je pense que nous pouvons et nous devons réussir, d'une part en relevant le niveau général, ça demande des efforts, ça demande du travail ça demande d'insister sur les matières fondamentales, en particulier le Français, les mathématiques mais aussi en relevant le défi de la mixité sociale et scolaire. Merci monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Lozach. Pour le groupe socialiste pour 2 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous le constatons depuis plusieurs décennies, notre système scolaire demeure profondément ségréguées. La corrélation entre le milieu socio-économique et la performance scolaire est l'une des plus fortes de l'ensemble des pays de l'OCDE, selon l'évaluation Pisa et elle s'aggrave chaque année sans que nous ne sachions y remédier. Qu'elle soit spatiale budgétaire résidentielle culturel cette segmentation sociale renforce les inégalités d'éducation et d'apprentissage nourri un sentiment de fatalisme et freine l'interaction entre élèves de différents niveaux. Les effets produits sont sévères et durables et participe à fracturer notre modèle républicain. Le code de l'éducation dispose que la scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Notre responsabilité et celle de votre ministère en particulier et de permettre à la Russie de tous les élèves, objectif fixé par la loi en améliorant partout les conditions de scolarisation en 1er lieu celle des plus fragiles. Aussi, Monsieur le Ministre, par quel moyen de lutter plus efficacement contre le séparatisme scolaire et contrer les stratégies d'évitement des familles. Comment développer une véritable culture de l'hétérogénéité dans les établissements. Sur des problématiques plus local qui impacte le fonctionnement de nos écoles et creuse plus encore les inégalités scolaires quand tant qu'entendez-vous opposé à la crise de structurelle du non-remplacement des enseignants dans nos départements qui dégrade les conditions d'apprentissage et sont à l'origine de fermeture de classe unique ou de sites isolés. Concrètement vous fermer des classes pour créer des postes de remplaçants. Exemple en Creuse dans un contexte national de suppressions de postes pour 2023 moins 1117 comment garantissez-vous une présence enseignante au quotidien dans chaque classe. Par ailleurs, la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers vous pas arrêter satisfaisante. Nous constatons sur le terrain de grandes difficultés dans la structuration et la complétude de nos Rased avec des zones blanches qui demeure enfin l'école du futur prônée par l'exécutif permettra-t-elle de réduire les inégalités territoriales telles que nous les subissons en hyper-ruralité ce dispositif vous paraît-il adapté à nos réalités. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur. Nous. La question du de l'évitement et du séparatisme scolaire dont vous parlez. Nous la pensons je la pense d'une double manière par le fait de rendre. Des établissements publics peu attractive de les rendre plus attractif. Nous en avons déjà parlé et également de faire de telle sorte que les établissements très attractif que les établissements favorisés, qu'ils soient publics ou privés s'ouvre et être une part d'élèves défavorisés plus importante si l'ensemble des propositions que j'ai fait ce soir. En ce qui concerne un point très important, c'est celui. De l'attractivité du métier d'enseignant, parce que, en effet, nous avons une question grave qui est celle de la perte d'attractivité du métier d'enseignant d'un rendement des concours qui est relativement faible de 83%. Ça veut dire que pour 100 postes mis au concours, on recrute 83 professeur. Ce qui fait d'ailleurs que la question. Du nombre de postes et de la baisse des moyens, elle doit aussi s'apprécier à l'aune du fait que ces postes ne sont pas toujours pourvu et donc. Avant de savoir s'il faut multiplier et augmenter le nombre de postes, il faut quand même aussi se demander si on arrive à mettre des professeurs dans les postes concernés. Donc la question de l'attractivité du métier est une question essentielle. C'est pourquoi il faut à la fois travailler sur l'augmentation des rémunérations car nos professeurs ne sont pas suffisamment rémunérés et nous faisons des propositions, j'ai nous sommes en négociation avec les organisations syndicales pour une part d'augmentation non conditionnelle de la rémunération des enseignants tous les enseignants. Des néo-titulaires jusqu'au dernier jour d'enseignement jusqu'à la retraite et puis une part conditionnel lié à de nouvelles missions, le tout pouvant représenter des augmentations substantielles mais je reconnais aussi que la question de l'attractivité du métier ne se résout pas seulement Le la rémunération il y a d'autres facteurs les carrières les déroulements de carrière, l'entrée dans le métier, les mutations les affectations tout cela. Nous y réfléchissons et nous allons faire des propositions dans les mois à venir pour faire de telle sorte que les postes soient pourvus, y compris dans les zones rurales. Merci, monsieur le Ministre. La parole est à madame Toine. Pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre, la mixité sociale est à l'école publique ce que les droits de l'homme sont pour la France une part de son être le résultat d'une histoire d'une politique de longue haleine. La première égalité c'est celle de l'accès au savoir. C'est le droit fondamental et inaliénable à une instruction que notre école publique n'était hélas plus en mesure de fournir à tous les enfants de notre pays. La crise de confiance qui pousse de plus en plus de parents se tourner vers le privé n'est pas le fruit d'une volonté, mais bien souvent une contrainte qui vise à contourner les failles de l'école publique. Le constat et les chiffres sont hélas connus dégradation du climat scolaire identifié dans un rapport du Sénat pointant le phénomène, pas de vague. Étiolement de l'autorité du à une politique du laisser-faire. Ajoutez à cela l'absence de reconnaissance d'un statut qui perd en attractivité vous obtenez logiquement une crise des vocations dans l'enseignement. C'est ce cocktail explosif qui empêche vraiment la mixité sociale. Laisser l'école publique se dégrader conduit mécaniquement à un déport vers le privé. Pour assurer une mixité sociale dans l'école de la République. Encore faut-il que le niveau général de l'instruction prodigué aux élèves soit redressé partout pour tous et dans la durée. Vous proposez de colmater un bateau dont il faut redresser le gouvernail par des bidons d'établissement un charcutage du car scolaire indigne des enjeux. Ne nous trompons pas de débat et encore moins de solutions. Monsieur le Ministre. Le sociologue Jean-Pierre Terrail rappelait en 2006 que les enfants de toutes les classes sociales peuvent mener une scolarité égal dès lors que le savoir transmis est le même partout. La maîtrise des acquisitions élémentaires neutralisent le poids de l'origine sociale dans les parcours scolaires là et donc la clé si l'on veut vraiment et durablement gommer le poids des inégalités sociales, comme l'a dit votre illustres prédécesseurs, Jules Ferry avec l'inégalité d'éducation je vous défie d'avoir jamais l'égalité des droits. Comment comptez-vous agir pour garantir à nouveau cette égalité et rétablir la mission essentielle et première de l'école publique. Je vous remercie. Merci monsieur le président, madame la sénatrice bourrin. Loin de moi l'idée de mettre en accusation qui que ce soit. En ce qui concerne. La mixité sociale et scolaire de chantiers importants le 1er et je vous rejoins ici c'est qu'il faut. Valoriser redresser dans certaines dimensions l'école publique. C'est pour cela d'ailleurs que nous poursuivons, ce qui a été engagé ces dernières années par exemple, le dédoublement. Des. Classes de grande section, CP, CE1 en éducation prioritaire. Il est presque achevée du côté des grandes sections des écoles maternelles. Nous poursuivons avec les plans français et mathématiques ou à l'école primaire avec la réforme du cours moyen l'insistance mise sur l'écriture. L'heure dégagé pour l'approfondissement et le soutien en français et mathématiques en 6e, ce sont des éléments substantiels, nous allons créer des clubs des mathématiques en grand nombre dans les collèges et dans les lycées avec Hugo Duminil-Copin notre médaille Fields. Nous avons réintroduit lors de mathématiques en première. Nous introduisons aussi des modules de renforcement en mathématiques en classe de seconde. Tout cela est fait pour valoriser solidifier l'école publique. À quoi j'ajoute des programmes spécifiques et les filières d'excellence. Nous en avons déjà parlé mais. La question de la sectorisation, madame la sénatrice, ça n'est pas du charcutage la sectorisation, ça se fait depuis toujours d'ailleurs et il est normal de penser la question de la sectorisation, en essayant d'obtenir. Les meilleurs résultats possibles. Les meilleurs résultats possibles. C'est des résultats. des résultats. Favorables pour les enfants favoriser bien entendu mais aussi des résultats qui fasse que les enfants défavorisés soit. Soit poussé en avant et c'est dans les établissements mixtes qu'on obtient ce type de résultats travaille sur le public mais aussi travaille sur la sectorisation et puis enfin, comme je l'ai déjà indiqué, participation de l'enseignement privé sous contrat. Nous faisons feu de tout bois pour améliorer les résultats scolaires de tous nos élèves. Merci. Ce Ministre monsieur Jacques Grosperrin. Pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci président, Monsieur le Ministre, un des objectifs de l'école et transmettre et de faire partager les valeurs de la République. La mixité sociale bien sûr doit y concourir, il favorise l'équité autorisé le meilleur pour la France des élèves mais toute la question est dans quelle condition mais 39 cet objectif. Il existe une tension majeure, le lien entre l'origine familiale et sociale et la composition sociale de l'établissement fréquenté. L'objectif se confronte à des résistants de tous les acteurs et ses actes. Ces indicateurs sont insuffisants. Avec une évaluation difficile et il est illusoire de prétendre analyser l'impact d'une seule variable dans l'ensemble de processus complexe les effets des égalités sont toujours comme il Le besoin exprimé fort il participe à la démocratisation de l'enseignement Clément anticipation républicaine. L'État a un devoir, celui de l'intégration réussie de toutes les composantes de la nation et la sectorisation scolaire et la ségrégation spatiale sont des outils essentiels qui était entré en conflit avec l'intérêt des familles sachant qu'en démocratie on ne peut leur reprocher de tenter d'obtenir les meilleures chances d'une scolarisation réussi pour leurs enfants. Tout est question d'équilibre dans l'action de l'État politique d'éducation prioritaire, eu le mérite de pointer du doigt les inégalités sociales et culturelles. Alors reconnu le besoin d'homogénéiser les karité sociale des élèves de certains établissements. Il faudra du courage en tout cas tous les jours sur la laïcité. Des objectifs et des actions sont annoncés. Lesquelles notamment avec les collectivités locales pour agir sur les affectations ce que scolaires ainsi qu'avec l'enseignement privé sous contrat. Pouvez-vous nous préciser les modalités. Lorsque vous affirmez qu'chacun devrait appartenir ou apporter sa contribution à l'effort de la refonte de la carte de l'éducation prioritaire. Mais quelle forme d'effort je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre. En France, les inégalités de naissance sont mal corrigé ou insuffisamment corrigée par l'école de ce point de vue là, la France a une situation particulière, c'est que dans beaucoup de domaines Les familles défavorisées sont aidées, elles sont mieux aider que dans de très nombreux autres pays en revanche sur l'école on on réussit moins bien en comparaison avec d'autres pays de l'OCDE et donc c'est c'est bien sur ce point qu'il faut. Se pencher, parce que les pays qui ont les meilleurs résultats par exemple certains pays d'Europe du Nord ou bien au-delà de l'Europe d'ailleurs. Sont des pays où les Delta les écarts. Entre les élèves sont les plus réduit sont les pays où le où il y a une plus grande homogénéité. De résultats scolaires et des sociétés d'ailleurs qui sont des sociétés moins illégal que la nôtre et donc nous devons travailler sur cette question. J'ai indiqué que notre méthode était celle de la concertation avec les collectivités. Parce qu'il n'y a pas une recette à appliquer. En revanche nous avons des objectifs et nous aurons des objectifs chiffrés. Cela concerne aussi l'enseignement privé sous contrat. Ce ne sera pas un simple engagement un peu vague et je me réjouis d'ailleurs de ce que nos partenaires de l'enseignement privé sous contrat soit tout à fait disposé à s'engager sur des objectifs chiffrés. Nous avons absolument besoin de progresser en la matière mais cela concerne aussi, j'insiste sur ce point les établissements publics, les établissements publics favoriser sur lesquels nous avons plus la main. Bien entendu, en particulier avec la sectorisation. Il ne s'agit pas de procédure de manière violente et bien entendu, que nous devons agir en concertation et en débat et en et en échange avec les associations de parents d'élèves avec les familles mais nous devons progresser à un rythme qui soit perceptible et visible de manière à obtenir des résultats significatifs, dès la rentrée 2024.

donc sur 25 pays de l'OCDE et qui monte que les meilleurs systèmes scolaire ce sont ceux qui remplissent 3 critères vous en citerai que de. Mise à part mise en oeuvre indépendamment du contexte culturel le 1er c'est la question d'un système scolaire ne peut excéder celle de son corps enseignant. Le 2ème, l'amélioration de l'enseignement dans les classes produit des résultats donc on parlait de formation tout à l'heure et Max Brisson. Il faudra peut-être s'interroger sur ce qui se passe véritablement classe et avoir le courage de le dire, de le faire et de l'évaluer, je vous remercie. collègues. Ce ministre-maire. Monsieur le président, Monsieur le Sénateur Grosperrin je je pense que la question de la formation des enseignants est une question absolument décisive et j'ai indiqué tout à l'heure que la formation aux métier était objectivement trop courte. J'ai fait une proposition d'ailleurs qui. Doit être étudiée et évaluée d'ailleurs dans toutes ses dimensions qui consisterait à recruter les professeurs des écoles à bac plus 3 au lieu de bac plus 5, en assurant 2 années de formation deux années d'élèves professorat en quelque sorte ce qui. Reviendrait.

Repense aussi la question du professorat des écoles dans sa dimension, je dirais d'ascenseur social parce que l'accès à bac plus 3 et socialement plus juste que l'accès à bac plus cinq et donc c'est quelque chose que je souhaite pousser c'est une transformation assez profonde du recrutement des professeurs des écoles. Si Monsieur le Ministre, Monsieur opérant. Je pense que vous êtes si Monsieur le Ministre, vos encouragements de monsieur Max Brisson. Je pense que c'est une bonne c'est une pas une bonne opération en tout cas c'est une bonne idée. Moi je voudrais revenir quand même ça fait de longues années que tous les ministres, tous les ministères ont mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, beaucoup d'attention dans les enseignements et depuis de longues années. On se rend compte qu'à travers les différents tests que soient pizza que soit Tim ce que ça soit d'autres tests nous moins bosser. On n'ose pas dire le mot de mauvais élèves ont toujours du mal à progresser, et puis les meilleurs sont toujours le meilleur. Donc il y a une véritable difficulté par rapport à cela et je pense que au delà. Mon cette annonce qui est intéressant et en tout cas qui qui peut participer à une amélioration de mots des élèves doit être aussi compléter, il faudra revenir sur ce que je disais tout à l'heure peut-être aussi s'interroger dans l'évaluation parce que la formation des enseignants, c'est fondamental, mais nous on le voit bien, lorsqu'on agrégé. Je ne suis pas sûr que ce soit les agrégés qui travaillent le plus là je vais avoir le courage de dire les choses. On le voit parfois et souvent ça dire qu'à un moment donné il faudra pouvoir améliorer dans le cas de la formation continue. Oui j'ai le courage de dire les choses. Monsieur le Ministre, parce qu'à un moment donné être. En tout cas politique c'est pouvoir dire comment redonner. Il faut que on regarde véritablement à ce qui se passe dans la classe et puis qu'on encourage ben ce qui travaillent peut-être un peu plus que les autres. Merci la parole est à madame Corinne Imbert pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur Ministre, chers collègues, nous le savons, en l'absence de mixité sociale à l'école, état des nombreux éléments préjudiciables à l'unité d'une nation. Si la question semble Seb, les réponses à apporter sont bien plus complexe opposant souvent et guide égalitarisme intransigeant et libertés individuelles. Ce mini-. Je ne vais pas abordé la question de la mixité sociale à l'école comme vous pourriez les vous y attendent ce sujet appelle nécessairement la question du mérite. Le mérite se par ce qui rend une personne digne d'estime de récompenses historiquement l'école républicaine permet à ses meilleurs éléments de s'élever dans la société. À force de travail et d'abnégation. Malheureusement ces dernières années ont été marquées par l'importation de des de débats venus d'outre-Atlantique. Fini l'universalisme républicain, place à l'assignation perpétuel dérivé du wokisme, le mérite n'existe plus car le monde se divise désormais entre oppresseur et oppressée catégorie orchestré en fonction de son jour de sa couleur de peau de son statut social et son orientation sexuelle. Votre seul mérite est alors aux yeux de ses théoriciens d'être dans le camp des victimes de l'oppression. C'est pas la même notion de de mérite. Ma question sera donc ça monsieur le ministre. À quoi bon louer certaines formes de mixité quand en même temps, on ferme les yeux sur l'apparition de nouveaux essentialiste racialiste au sommet d'une de l'éducation nationale qui, sous couvert de lutte quand toutes les formes de discrimination enferme les individus dans des stéréotypes qui compromettent l'équilibre même de notre pacte républicain, je vous remercie. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Imbert. La notion de mérite j'y souscris entièrement quant à penser que l'école jadis. Aurait été l'école du mérite pour tous. J'ai indiqué précédemment qu'il fallait regarder d'un peu plus près. Tant l'école de jadis justement était une école inégalitaire, l'école de Ferry. L'été pensé pour éduquer les enfants du peuple. Les enfants de la paysannerie comme les enfants du monde ouvrier, mais jusqu'au certificat d'études, quelles que soient les mérites des enfants concernés. Le pourcentage d'élèves qui avaient le bac au début du XXe siècle c'était quelque chose comme un pour 100 de la population, on est évidemment dans un monde que. Particulièrement inégal et particulièrement lié. Aux positions sociale. Des familles. Les lycées étaient réservés à une minorité bourgeoise et je rappelle à cet égard que les instituteurs du début du XXe siècle n'allait pas au lycée. Et il n'obtenait pas d'ailleurs le Baccalauréat puisqu'ils entraient dans les écoles normales qui était une filière conçu justement pour élever jusqu'au jusqu'aux instituteurs justement jusqu'au métier d'instituteur. Les enfants du peuple. Donc je n'ai pas de nostalgie particulière pour une époque qui était une époque très inégalitaire. Je ne suis pas sûr de voir ce que vous voulez. dans la situation de l'école d'aujourd'hui dans une école qui serait une école wokistes. Si je comprends bien, je demande à regarder et regarder avec moi les programmes. D'histoire, de géographie de SVT, les programmes de l'être. Je ne vois pas très bien en lisant ses programmes en lisant les instructions pédagogiques et en regardant ce que font les enseignants. Je ne reconnais pas. Le dans tout cela. Le, le tableau que vous tracez. Merci, monsieur le Ministre Madame Aubert. vous avez dit que vous étiez attachés. Je n'ai pas le le le regret de l'école d'autrefois. Néanmoins je ne comparerai pas. Le bac d'aujourd'hui et le certificat d'études des personnes n'ont eu que leur certificat d'études étaient pour autant des personnes très intelligente et vous l'avez dit vous-même la formation des instituteurs d'autrefois même sur le Baccalauréat conduisait à à des hommes et des femmes. Je crois digne bien éduquées et capables de transmettre leur savoir et très attachés à leur métier. Alors le le débat sur l'autre qui souhaite effectivement un autre débat, mais je voulais l'introduire, parce que c'est une façon aussi à la fois de de fracture sociale et. Renvoyé peut être à des déclarations dans 12 d'autres domaines, vous preniez des réunions en non-mixité alors qu'aujourd'hui on parle de mixité sociale à laquelle je crois aussi pour plus d'égalité. Je vous remercie. Madame Béatrice Gosselin pour le groupe puis qui tient pour 2 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Toutes les enquêtes concordent. La France est l'un des pays où le milieu social de l'élève conditionne le plus sa réussite scolaire. Cette situation n'évolue pas. Malgré les réformes qui se sont succédé ces dernières années. Pour assurer l'égalité des chances. Monsieur le Ministre, vous comptez agir sur la mixité sociale principalement au collège et au lycée. Mais le sort de l'élève se joue bien avant. Selon les données de l'de l'Institut national d'études démographiques en début de CP, seuls 42% des élèves inscrits dans les dans les écoles en REP plus ont une bonne compréhension du de la de la langue à l'oral. Les 75% des écoles, des élèves des écoles situées hors de ses territoires. 46% des premiers ont un niveau satisfaisant résolution de problèmes mathématiques, contre 70% pour les seconds. L'observe l'Observatoire des inégalités, relève que déjà à la maternelle les tout petits ont tu ne maîtrise inégale du vocabulaire les enfants issus de l'immigration, notamment de peuvent progresser au même rythme que ceux d'une famille aisée. Or ce sont pendant les premières années de son existence que l'enfant dispose des meilleures capacités cognitives pour l'acquisition du langage et du raisonnement. Ma question porte donc sur la nécessité d'intervenir le plus tôt possible dans l'éducation des jeunes élèves issus d'un milieu modeste. Monsieur le Ministre, vous avez annoncé un plan pour les maternelles. Sans préciser quelles mesures concrètes seront prises et les moyens dont vous disposez. Je rappelle que de nombreuses classes de maternelle sont en sureffectif et que le nombre de postes d'Atsem et d'AESH accompagnants les enfants est toujours insuffisant. Pourriez-vous nous apporter des précisions concernant vos projets pour cette période déterminante. Je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Gosselin. La question de la mixité sociale et scolaire se pose effectivement plus dans, au collège et au lycée. Ça ne veut, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas s'intéressent Aux primaires, que ce soit. Aux écoles maternelles ou aux écoles élémentaires. Je rappelle à cet égard les efforts réalisés ces dernières années en matière de dédoublement en éducation prioritaire pour les grandes sections pour les CP et les CE1. Les résultats des premières cohortes entré en dents ayant bénéficié de ces dédoublements et qui sont désormais en en sixième. Nous avons les évaluations de 6ème qui indique Des progrès intéressants en ce qui concerne surtout les enfants de REP plus. Des progrès qui ont été cependant embarrassée ou en tout cas entravée par la crise sanitaire, avec le confinement dont nous n'avons pas fini de payer les conséquences, à tous égards, que ce soit sur la santé psychique et physique des enfants mais aussi sur leur niveau scolaire. Par ailleurs, donc nous poursuivons le dédoublement il nous achevons nous sommes à environ à 75% pour les 2 doublement des grandes sections, notre objectif c'est de parvenir à 100%. Ans pour la rentrée 2024. Par ailleurs. Vous savez, nous sommes favorables en ce qui concerne l'éducation prioritaire à l'ouverture de toute petite c'est de très petite section à la scolarisation des enfants avant 3 ans, qui donne de bons résultats, notamment pour ce qui concerne l'acquisition du vocabulaire et j'ai pu moi-même visiter des très petites sections dans des écoles maternelles de quartiers prioritaires dans le Sud-Ouest de la France. Pour ce qui concerne le plan maternelle celui-ci à plusieurs volets, un volet notamment de formation des enseignants de maternelle puisque les enseignants. Du les professeurs des écoles sont globalement formés de la même manière que ce soit les enseignants de maternelle de petite section où les enseignants de CM2. Il paraît intéressant, utile, surtout en comparaison d'autres pays de. Spécial sinon de spécialisée en tout cas d'apporter des compléments de formation. Aux enseignants. Des écoles maternelles. Le plan maternelle a une dimension importante relative aux fonctions au à la formation des enseignants de maternelle. Merci Madame Gosselin. Oui, monsieur le Ministre quand vous dites que vous que le Covid a fait des dégâts au niveau de nos enfants, c'est vrai, mais quand on voit combien de classes sont fermées. Cette année, dans un département comme la Manche, où on a fermé 9 classes. L'an dernier pour 380 élèves en moins et que cette année pour 550 élèves en moins on enferme 3 29, je vous assure qu'on est inquiet sur le devenir de nos et de nos enfants. Merci. Merci. Donc pour conclure ce débat. La parole est à madame madame Sylvie Robert pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour cinq minutes. Oui merci merci Monsieur Président. Alors en conclusion de ce débat, d'abord je voudrais remercier les les collègues qui par leurs différentes interventions et leurs points de vue ont vraiment témoigné de leur intérêt pour. Pour cette question de, de la mixité scolaire, scolaire. Je voudrais également remercier le ministre. À la fois bien sûr pour ses réponses toujours étayer mais aussi pour les quelques annonce. Qu'il a pu nous faire et je trouve important. Que vous ayez dans la suite de votre réflexion sur cette question qui est aujourd'hui pour moi en tout cas que je qualifie d'enjeu démocratique et la publication des IPS nous engage, on peut le dire comme ça et et cette réalité là en tout cas elle ne peut que nous inciter à aller plus loin. Hé bien que ces annonces que vous avez fait en tout cas que ce que vous nous avez dit vouloir pousser comme vous dites, par la négociation par le temps et bien. Et nous puissions en en tout cas. Avec vous et et en tout cas au Sénat parce que vous avez vu qu'il y a un intérêt réel pour cette question. Hé bien pouvoir en tout cas en avoir. dans dans les dans les semaines à venir. Alors c'est vrai que par les interventions. Les collègues ont beaucoup et vous évoquez les moyens parce que au-delà de la question de la mixité scolaire, vous avez tous tous évoqué la question des des des moyens et et Béatrice Gosselin bien vient de le faire d'ailleurs à travers, à travers ses propos mais on a bien vu aussi que pour cette question là. Les leviers sont multiples et et et on on a pu en évoquer certains vous l'avez monsieur Ministre aussi évoqué la qui sont des options, la question des des des différents parrainage en tout cas des. tout ça la sectorisation. Je crois que les leviers sont sont multiples et que il va falloir vraiment pouvoir tenter de les actionner parce que derrière cela il y a aussi de l'interministériel, la politique de l'habitat, de l'aménagement du territoire de la Fabrique de nos villes et de nos territoires. Que ce soit en milieu en milieu rural ou en milieu urbain parce que la question de la ruralité aussi vous l'avez évoqué et des spécificités. Je pense que ça, il faut absolument vraiment le souligner le partenariat avec les collectivités forcément mais aussi la formation des enseignants et à cet égard et pas seulement sur la formation des 100 seniors mais puisqu'on voit bien que c'est une palette, vous l'avez dit vous-même extrêmement diverses. Eh bien comme on a beaucoup parlé d'expérimentation de la Haute-Garonne. Moi j'encourage les collègues. qui ce qu'il en a été fait, c'est-à-dire le rapport qui a été rendu aux deux, je crois que c'est 4 ans 5 ans d'expérimentation parce qu'on voit bien que d'abord ça a donné des résultats comme on l'a dit extrêmement positif mais que cette expérimentation a été aussi l'occasion d'actionner tous ces leviers tous ces leviers et ça et je l'ai dit dans dans dans mes propos liminaire, ça demande aussi des moyens. Et, et je crois que je reviens aux moyens budgétaires mais ça peut être en tout cas l'occasion de de de pouvoir. Eh bien travailler au plus près avec les, les collectivités territoriales sur peut être leur volonté d'expérimenter d'autres d'autres projets de cette nature. Alors pour terminer parce que je, je ne veux pas être trop longue. Vous nous avez parlé du 20 mars. On a beaucoup parlé des de l'école privée sous contrat puisque cette question qui arrive dans notre débat quand même pour travailler sur l'amélioration de la mixité scolaire. Vous avez dit être en négociation aujourd'hui et que vous nous donneriez peut être en tout cas la teneur d'un protocole d'accord qu'il arriverait aux alentours du 20 mars. Je pense que nous sommes très impatients à voir et regarder ce qu'il contient. Parce que derrière cela il y aura aussi forcément je dirais peut être une autre étape. Dans ce XXIe siècles sur cette question de, de, de mixité scolaire, je crois vraiment et je terminerai par là pour vous dire que et on le voit dans d'autres pays, c'est véritablement un enjeu démocratique et républicain, et je crois que c'est une promesse que l'on doit tous les enfants de notre pays et que pour cela il faut il faut un grand volontarisme politique en tout cas, on compte sur vous Monsieur le Ministre, merci. Merci. Mes chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance ce jeudi de mars à 10h 30 pour les questions orales. La séance est levée.